La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du lundi 2 octobre a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. j'ai reçu les déclarations des présidents de groupe qui souhaitent être reconnus comme groupes minoritaires ou groupes d'opposition au sens de l'article 51-1 de la Constitution. M. Didier Guillaume, président du groupe socialiste et républicain, et Mme Éliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ont fait connaître que leurs groupes se déclarent comme groupes d'opposition. M. Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste, M. François Patriat, président du groupe La République en marche, M. Jean-Claude Requier, président du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, M. Claude Malhuret, président du groupe République et Territoires/Les Indépendants, ont quant à eux fait savoir que leurs groupes se déclarent comme groupes minoritaires. Chacun de ces groupes pourra donc, au cours de la session, bénéficier des droits attribués aux groupes d'opposition et minoritaires par la Constitution et notre règlement, notamment dans le cadre des « espaces » qui leur sont réservés. L'ordre du jour appelle la désignation des vice-présidents, questeurs et secrétaires du Sénat et la proclamation de la constitution du bureau définitif. Conformément à l'article 3 du règlement, la liste des candidats à chacune de ces fonctions a été publiée à douze Cette liste n'a fait l'objet d'aucune opposition pendant le délai réglementaire. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame vice-présidents MM. Philippe Dallier, David Assouline, Mme Valérie Létard, MM. Jean-Marc Gabouty, Thani Mohamed Soilihi,

Je proclame secrétaires M. Éric Bocquet, Mme Agnès Canayer, M. Yves Daudigny,

Mme Patricia Schillinger remplacera Mme Mireille Jouve en qualité de secrétaire du Sénat à compter du 1 avril 2019 à zéro heure. Je déclare le bureau du Sénat constitué. Communication en sera donnée à M. le Président de la République, à M. le Premier ministre et à M. le président de l'Assemblée nationale. Je félicite chacun des membres du bureau du Sénat qui, je les en assure déjà, ne manqueront pas de travail, qu'ils soient vice-présidents, questeurs ou secrétaires ! Je vais

aux sept commissions permanentes et à la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne, et de leur ratification sauf opposition dans le délai d'une heure.